J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer des textes sur les dispositions restant en discussion des projets de loi organique et ordinaire relatifs à la dette sociale et à l'autonomie ne sont pas parvenues à l'adoption de textes communs. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Viviane Artigalas.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la transposition de directives européennes dans notre droit ne peut être prise à la légère malgré sa grande technicité. Elle demande une attention particulière de la part du Parlement. Or, en la matière, je ne peux que rappeler, comme l'ont déjà fait mes collègues, les conditions de travail qui ont présidé à l'examen de ce texte. Ce projet de loi a été présenté en conseil des ministres le 12 février dernier, alors qu'il devenait urgent pour la France, qui assurera à partir du 1 janvier 2022 la présidence de l'Union européenne, de n'afficher aucun déficit de transposition. Malheureusement, son examen intervient dans un contexte particulièrement tendu d'après covid-19. On peut donc regretter de devoir une fois de plus travailler dans l'urgence et par le biais d'habilitations à légiférer par ordonnance sur des sujets qui constituent des enjeux politiques complexes nécessitant l'avis du Parlement, alors que ce texte aurait pu être travaillé dès l'automne 2018.

Malgré ces difficultés de forme, sur le fond, ce texte apparaît comme globalement positif, car il permet la transposition de nombreuses dispositions très attendues. Les dispositions relatives à la protection des consommateurs renforcent la lutte contre les mauvaises pratiques de commerce en ligne, notamment face aux sites frauduleux, et rendent obligatoire la garantie de conformité pour les biens et données numériques. Elles obligent également les plateformes numériques à répondre à un certain nombre d'exigences en matière de transparence et de loyauté. Quatre directives- contre les pratiques commerciales déloyales, relatives aux droits des consommateurs, aux clauses abusives dans les contrats ou encore à l'indication des prix -imposent de nouvelles règles d'information et d'encadrement des pratiques. Les dispositions relatives à la lutte contre le blocage géographique injustifié au sein du marché intérieur et, surtout, sur le territoire national étaient particulièrement souhaitables. En effet, il était anormal que persistent certaines pratiques discriminatoires envers les consommateurs, en raison par exemple de leur lieu de résidence. Concrètement, ces directives empêcheront que des utilisateurs voient leur accès à un site internet ou à une application développés dans un autre État membre limité pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu de connexion de l'ordinateur. Ces dispositions restent importantes pour nos concitoyens, en particulier pour ceux des outre-mer. Pour autant, les États membres ne sauraient faire l'économie d'un véritable plan de régulation du numérique qui garantira la liberté de choix des internautes et les protégera en tant que citoyens et consommateurs, notamment face à la montée en puissance des Gafam et de leur équivalent chinois. C'était tout le sens des travaux rendus par la commission d'enquête sénatoriale sur la souveraineté numérique, qui préconisait de définir une véritable loi d'orientation et de suivi et d'user des leviers du multilatéralisme pour encourager les innovations au niveau européen. Les dispositions relatives à la zootechnie et à la santé animale appellent peu de commentaires, tant il est vrai que les États disposent de peu de marge de manoeuvre pour transposer ces règlements hypertechniques. À ce stade, nous savons fort peu de choses et nous ignorons les intentions du Gouvernement sur le fond. Nous estimons donc que le projet de loi de ratification nécessitera une vigilance accrue du Parlement. Enfin, je tiens à saluer la décision de la commission des finances, qui a adopté les amendements concordants du rapporteur et du groupe socialiste visant à supprimer l'article 23 relatif au Brexit et la moitié de l'article 24 relatif à la répartition future des compétences entre l'État et les régions sur la gestion du Feader. Dans ce cas précis, il est totalement anormal que le Gouvernement utilise un projet de loi de transposition pour aborder la question des compétences des régions sans aucun débat ni consultation préalable. Est-ce par le biais d'ordonnances que l'État entend traiter un sujet aussi sensible que celui de la décentralisation Contrairement aux conclusions de l'étude d'impact du projet de loi, certaines régions, comme l'Occitanie ou la Nouvelle-Aquitaine, s'opposent à la volonté du Gouvernement de retirer totalement aux régions la responsabilité des mesures surfaciques- ICHN, soutien à l'agriculture biologique et mesures agroenvironnementales et climatiques liées à la surface. Il est donc faux de dire que les principaux acteurs concernés y sont favorables. J'ose espérer, monsieur le ministre, qu'un sujet aussi crucial pour l'équilibre de nos territoires fera l'objet d'un véritable débat parlementaire, et non d'un examen au détour d'un projet de loi dont l'objet en reste assez éloigné. En tout état de cause et malgré les difficultés que j'ai soulignées, nous voterons ce projet de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'Union européenne se construit et se consolide souvent en période de crise- celle que nous traversons le démontre encore. Mais l'Europe agit aussi au quotidien pour améliorer la vie de nos concitoyens. Cette facette de la politique européenne n'est pas toujours suffisamment perceptible. Ce texte nous donne l'occasion Le projet de loi que nous examinons a pour objectif de traduire dans le droit national les avancées issues de la réglementation européenne. Dans ce projet de loi de vingt-quatre on ne dénombre pas moins de quatorze demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance. La commission, pourtant très vigilante quant au recours aux ordonnances, a laissé dans le texte une grande majorité de ces demandes d'habilitation tout en réduisant leur nombre.

les domaines très divers traités dans ce texte, l'agroalimentaire me tient particulièrement à coeur, car, y compris au sein de l'Union, les relations commerciales entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs demeurent déséquilibrées, trop souvent aux dépens des agriculteurs et des PME. Il est donc nécessaire de fixer des règles communes pour des relations commerciales plus saines, plus équilibrées. Ce texte permet de rétablir et de garantir la loyauté de transactions commerciales dans la chaîne alimentaire. La transposition des règles européennes en matière de lutte contre les maladies animales est également nécessaire. Nous avons besoin d'un cadre juridique harmonisé pour permettre à nos éleveurs de participer plus équitablement au jeu de la concurrence sur le marché européen. Il faut dire que les éleveurs français font face à une réglementation sanitaire des plus exigeantes. C'est une garantie pour nos consommateurs, mais cette qualité a nécessairement un coût pour les éleveurs. Il faut donc en faire un atout à valoriser et, bien évidemment, à harmoniser. À cet égard, je me réjouis que nous conservions notre avance concernant le suivi des maladies animales. C'est une exigence de qualité et une garantie pour nos éleveurs. Je partage également pleinement les propositions portées par la commission sur la surveillance des

nous ont rappelé l'importance des enjeux de veille sanitaire. L'Union européenne est donc une source majeure de progrès pour les Européens. Ses avancées sont sans doute discrètes mais multiples et ô combien concrètes sur nos territoires pour le quotidien de nos concitoyens. Le groupe Les Indépendants votera ce texte enrichi par les travaux des commissions et des rapporteurs ainsi que par le débat parlementaire. La parole est à M. Jean-Pierre Leleux. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais évoquer ici un sujet qui s'est invité dans l'examen du présent texte : la protection de la création audiovisuelle française et de nos auteurs. En effet, le Gouvernement a souhaité introduire dans le projet de loi par voie d'amendement la transposition de trois importantes directives européennes. La première est la directive Services de médias audiovisuels, dite SMA, du 14 novembre 2018, dont la transposition est urgente puisqu'elle doit avoir lieu avant le 19 septembre 2020. Nous avons tous à l'esprit

Lors des négociations, la France a joué un rôle majeur pour imposer le respect de notre modèle de financement de la création. Dans la même logique, la directive prévoit des mesures visant à rompre avec l'asymétrie des situations entre anciens et nouveaux acteurs de l'audiovisuel, par exemple en autorisant le placement de produits. Elle permet également d'actualiser les compétences de l'instance de régulation- actuellement, le CSA -, notamment en ce qui concerne le contrôle des plateformes de vidéo à la demande. La deuxième directive destinée à être transposée est la directive dite Droit d'auteur du 17 avril 2019. Après deux années de vifs débats, l'Union européenne a validé le principe d'une meilleure rémunération des artistes et éditeurs de presse à l'occasion de la diffusion de leurs contenus sur des plateformes comme Google ou YouTube. Assurer le respect des droits d'auteur sur les plateformes s'est avéré compliqué dans la mesure où les oeuvres sont téléversées par les utilisateurs des services de partage et non par les services eux-mêmes. La directive européenne rend finalement les plateformes responsables des contenus publiés et les oblige à conclure des accords avec les ayants droit des oeuvres pour qu'ils soient rémunérés ou à retirer les contenus dont la publication ne respecterait pas le droit d'auteur.

qui franchit une étape supplémentaire en faveur de la modernisation du droit d'auteur en Europe en facilitant la cession de droits pour les services de radiodiffusion par satellite et de retransmission par câble sur le marché unique de l'Union européenne. Le présent projet de loi, parce qu'il vise à transposer plusieurs réformes importantes récemment introduites dans la législation de l'Union européenne, peut devenir, en raison de circonstances exceptionnelles, le véhicule de transposition de ces trois directives. la transposition des directives devait être assurée par l'adoption du projet de loi pour une réforme de l'audiovisuel, mais, nous le savons, l'examen de celui-ci s'est trouvé brutalement interrompu à l'Assemblée nationale au moment de la crise sanitaire. Or l'ensemble des professionnels concernés attendent cette nouvelle règle.

que cette procédure a déjà été fort utilisée lors de l'état d'urgence et que, en l'espèce, le Gouvernement est largement responsable du présent retard de transposition, le calendrier de la réforme audiovisuelle ayant été sans cesse reporté depuis

dans un calendrier déjà très chargé. L'adoption de ces dispositions par le Sénat permettrait leur promulgation fin juillet. Ensuite, comme je l'ai expliqué, ces directives contribuent à réaffirmer notre souveraineté culturelle à l'ère numérique, à permettre la rémunération de nos auteurs et à faire participer les acteurs étrangers au financement de notre création. Or les acteurs français de l'audiovisuel et de la création ont d'autant plus besoin d'aide que les circuits de financement ont été gravement fragilisés par la crise sanitaire- je pense notamment à la chute des recettes publicitaires -alors que les plateformes, au contraire, ont pu augmenter leur chiffre d'affaires. Enfin, la France, qui a toujours été pionnière sur ces sujets, serait le premier pays européen à assurer la transposition des directives, permettant aux autres pays de reprendre tout ou partie de sa rédaction. Encore faut-il se garder d'une transcription trop rapide qui ne respecterait pas l'équilibre recherché par le projet de loi Audiovisuel entre les plateformes, d'une part, et les acteurs nationaux, d'autre part. Lors des auditions menées par le groupe de travail Médias audiovisuels au sein de notre commission de la culture, nous avons pu constater la déception des chaînes françaises face à la méthode retenue par le Gouvernement. En effet, la directive SMA intègre les plateformes dans le système de financement de la création française, mais il ne faut pas oublier que cette mesure devait avoir pour corollaire l'assouplissement des obligations pour les acteurs historiques. Or si le calendrier de la transcription de la directive est maintenant accéléré, votre prédécesseur, madame la ministre, avait renvoyé à une date ultérieure indéterminée les aménagements pour ces acteurs traditionnels. Les éditeurs de programmes nous ont fait part de leurs inquiétudes, car les nouvelles productions locales, financées par les plateformes, auront pour effet paradoxal de renforcer leur attractivité, avec des productions premium sur lesquelles elles auront des droits élargis. Si la directive SMA est une bonne nouvelle pour les producteurs, elle risque d'accroître l'écart entre les nouveaux acteurs et les anciens,

dans la réglementation appliquée aux différents acteurs afin d'assurer, à l'avenir, des conditions de concurrence plus justes. Je présenterai en ce sens un sous-amendement à l'amendement du Gouvernement relatif à la directive SMA afin d'introduire dans le texte ce principe d'équité. Madame la ministre, monsieur le ministre, dans un temps réduit un dialogue constructif avec vos services sur cette idée d'équité- je salue la qualité de nos échanges. L'introduction du principe d'équité constitue un symbole politique fort, puisqu'il signifie que le Gouvernement devra veiller à rétablir à rétablir des conditions de concurrence plus justes entre les acteurs historiques, dont les obligations ont été définies il y a plus de trente ans dans un univers fermé sans concurrence internationale. Ce principe aura également une portée juridique, puisqu'il s'imposera en particulier au pouvoir réglementaire et devra donc s'appliquer dans les mois à venir. L'adoption par notre groupe de dispositions transposant cette directive sera conditionnée à l'adoption de ce sous-amendement issu des travaux de notre groupe de travail. Ce n'est pas seulement l'avenir de l'économie du secteur, mais également celui de l'exception culturelle française qu'il s'agit ainsi de préserver. Très bien

de transcrire cette directive en droit français. Le fait de la transcrire maintenant est plutôt positif, puisque

nous avons déjà eu l'occasion de débattre très longuement du sujet lors de l'examen de la proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace. Je ne m'attarderai Je ne m'attarderai donc pas sur le fond et rappellerai simplement que ce texte a pour objet d'éviter la domination excessive de quelques plateformes structurantes et la restriction de la liberté de choix des consommateurs qui en résulte.

ses propositions rejoignent d'ailleurs très largement les orientations définies dans notre proposition de loi -, mais ce n'est que le début d'un processus législatif européen qui, par nature, sera très long. Le Gouvernement sait bien qu'il existe des divergences entre les États membres sur le sujet et que l'adoption définitive d'un texte en la matière

l'interopérabilité des plateformes, la lutte contre les acquisitions prédatrices et l'encadrement des interfaces trompeuses ont été adoptées à l'unanimité par le Sénat. Monsieur le ministre, nous ne pouvons plus nous permettre d'entendre des arguments tendant à remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. L'épisode récent de l'application StopCovid l'a bien montré. Nous le voyons avec le présent projet de loi, le Gouvernement tarde trop souvent à transposer les textes européens

Il estime en revanche que ce constat appelle une autre réponse que celle qui est proposée. La nouvelle Commission européenne vient de prendre deux initiatives fortes et importantes.

La France a beaucoup plaidé et agi pour que l'Union européenne se dote de nouveaux instruments à la hauteur des enjeux et des défis de l'économie numérique. Elle continuera à travailler très étroitement avec ses partenaires européens, afin que cet objectif soit atteint aussi rapidement que possible. Nous avons besoin d'une Europe plus forte pour protéger les consommateurs et garantir le bon fonctionnement du marché face aux grands acteurs mondiaux du numérique. Les autorités nationales auront leur rôle à jouer dans le nouveau cadre que nous appelons de nos voeux, mais il est impératif que, face à ces acteurs mondiaux, les principes et l'architecture de la nouvelle régulation soient définis au niveau européen. Des initiatives nationales en ordre dispersé seraient de notre point de vue inefficaces : cela permettrait aux grands acteurs du numérique de jouer les États les uns contre les autres. Ce qu'il faut, c'est un marché intérieur européen renforcé et plus protecteur.

Cet amendement a été déposé à la suite d'une proposition de loi cosignée par de nombreux sénateurs socialistes. Il soulève la question de la régulation économique du numérique et de la liberté de choix des utilisateurs d'internet en tant que consommateurs et citoyens.

elle le rappelle aujourd'hui, « les mesures proposées ont vocation à constituer un dispositif pilote dans les négociations internationales et européennes sur ces sujets ». Encore une fois, monsieur le ministre,

l'interopérabilité pour obliger les plateformes à respecter un certain nombre de modes de régulation. Nous avons eu ce débat à plusieurs reprises. Je n'ai jamais entendu le Gouvernement dire, dans cet hémicycle, qu'il était favorable

Vous allez découvrir les travaux du Sénat- j'en profite pour vous féliciter de votre nomination. De longue date, nous travaillons sur les questions de souveraineté numérique, du pouvoir incommensurable des plateformes, qui se sont constituées en oligopoles qui empêchent tout développement à terme de notre économie, voire la menacent très fortement. On sait bien que c'est au niveau européen qu'il faut légiférer. Je vous renvoie au rapport fait

J'entends bien ce que l'ensemble des intervenants ont dit. La volonté du Gouvernement est de donner sa chance à une solution européenne, mais, vous avez raison, il ne faut pas traîner.

relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire comporte, pour partie, les dispositions figurant initialement dans l'article 5 du présent projet de loi. Toutefois, cet article ne reprend pas les mesures permettant à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de lutter efficacement contre les contenus illicites en ligne, qui figuraient initialement dans l'article 5. Il s'agit ici de lutter aussi bien contre les petits sites internet d'arnaques en tout genre, qui empoisonnent la vie de nos concitoyens, notamment ceux qui se font passer pour des sites de l'administration ou d'entreprises connues, que contre les places de marché qui laissent en ligne des produits représentant un danger pour la santé ou la sécurité alimentaire et non alimentaire des consommateurs. Le présent amendement vise à reconnaître à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation le pouvoir d'ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne, c'est-à-dire aux personnes qui exercent une activité de classement ou de référencement- les sites de comparateurs, les moteurs de recherche ou encore de mise en relation de plusieurs parties places de marché, mais aussi aux fournisseurs d'accès à internet ou à un navigateur l'affichage d'un message d'avertissement visant à informer les consommateurs du risque grave de préjudice pour leur intérêt que représente un contenu illicite en ligne. Pour les infractions les plus graves, cet amendement reconnaît à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation la possibilité- pouvoir B1 de déréférencement -d'enjoindre aux opérateurs de plateformes en ligne le déréférencement des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, ou d'enjoindre- pouvoir B2 de filtrage -aux différents acteurs précités, mais aussi aux simples hébergeurs d'en empêcher l'accès et- pouvoir B3 de blocage de noms de domaine -d'ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d'un nom de domaine. Ces mesures sont proportionnées à l'objectif de protection des consommateurs, car elles sont graduées. Elles ne seront mises en oeuvre que lorsqu'aucun autre moyen efficace n'est disponible pour faire cesser le manquement ou l'infraction, c'est-à-dire lorsque le responsable du contenu manifestement illicite ne peut être identifié ou qu'il n'a pas répondu à une injonction de cessation de la pratique en cause. Elles ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque la pratique est manifestement illicite. Les pouvoirs B ne peuvent être mis en oeuvre que pour les pratiques les plus graves, uniquement celles qui sont punies d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à deux années il existe un risque de préjudice grave pour les intérêts, notamment sanitaires, des consommateurs. Enfin, dans le cadre d'une procédure de transaction administrative, cet amendement a pour objet de permettre à l'administration de prononcer une sanction administrative

à M. le rapporteur pour avis. L'amendement du Gouvernement permet de concilier à la fois l'efficacité de l'action de la DGCCRF pour lutter contre les infractions qu'elle repère sur les sites en ligne et le respect des droits et libertés publiques. publiques. Dans la version initiale de l'article 5, le Gouvernement envisageait d'octroyer à la DGCCRF un pouvoir substantiel, qui était certes utile dans sa finalité, mais qui n'était assorti d'aucune garantie quant à l'atteinte au droit de propriété ou à la liberté du commerce et de l'industrie. Ce faisant, un tel dispositif présentait un risque majeur d'inconstitutionnalité. C'est la raison pour laquelle le Sénat avait adopté un amendement lors de l'examen du projet de loi portant

: il vise à mieux encadrer le nouveau pouvoir de la DGCCRF, qui sera gradué en fonction de la gravité des infractions commises et limité au contenu en ligne manifestement illicite, lorsque son auteur ne pourra être identifié ou qu'il n'aura pas déféré à une première injonction. Pour autant, il nous semble que la rédaction de cet amendement doit encore évoluer, afin de clarifier certaines incertitudes en ce qui concerne les types de manquements visés et les acteurs auxquels la DGCCRF pourra demander de réduire l'accès à des interfaces en ligne, dont les contenus sont manifestement illicites. Tel est l'objet du sous-amendement que je vous propose. Ce sous-amendement vise que les manquements et infractions concernés seront ceux qui enfreignent les règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits, ainsi que ceux qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs. à prévoir que les professionnels auxquels la DGCCRF pourra ordonner l'affichage d'un message d'avertissement seront les opérateurs de plateformes en ligne, les fournisseurs d'accès à internet, ainsi que les navigateurs. Ceux auxquels elle pourra notifier les adresses électroniques, afin qu'ils en limitent l'accès, seront les fournisseurs d'accès à internet, les navigateurs, les opérateurs de plateformes en ligne et les hébergeurs. Enfin, le présent sous-amendement a pour objet de préciser que, dans le cadre d'une transaction administrative, la DGCCRF ne pourra reprendre la procédure de sanction classique que dans le cas où

c'est-à-dire lorsque l'accord comporte des engagements de la part de la personne incriminée ou en cause, un litige né de son inexécution devra être

Un délai de neuf mois permettra de respecter l'échéance de transposition fixée par la directive, tout en procédant à une large consultation des professionnels, à laquelle le Gouvernement tient et s'est engagé, à l'instar des consultations menées à l'occasion de la refonte du compte de commerce en avril 2019.

qui, largement inspirée par le droit français des pratiques commerciales restrictives (PCR), constitue une avancée majeure pour l'harmonisation de la loyauté et de la transparence des relations interentreprises en Europe. De nombreuses pratiques commerciales qualifiées d'abusives par cette directive sont depuis longtemps prohibées en droit français, notamment la prohibition du déséquilibre significatif, de l'obtention d'avantages sans contrepartie ou de la rupture brutale des relations commerciales, et sont d'ores et déjà applicables à toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires annuel, le droit français des PCR étant de type « symétrique ». Toutefois, certaines d'entre elles ne le sont pas et doivent donc être transposées. Cependant, la directive impose une transposition de type « asymétrique » et sectoriel : elle demande de les interdire lorsqu'elles interviennent dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires d'un fournisseur avec un acheteur d'une plus grande taille et au chiffre d'affaires plus important. La commission du Sénat a supprimé la condition de chiffres d'affaires, optant ainsi pour une surtransposition et un dispositif de type « symétrique ». Cet élargissement à toutes les entreprises devrait cependant pouvoir être différencié en fonction du chiffre d'affaires des opérateurs concernés selon les pratiques prohibées par la directive, afin de rendre la réglementation plus pertinente, plus pragmatique et donc plus efficiente. Tel sera d'ailleurs l'objet d'une consultation des professionnels que le Gouvernement entend mener.

qui promeut l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, entre en vigueur le 12 juillet 2020. L'habilitation à mettre en oeuvre ce règlement par voie d'ordonnances n'est aujourd'hui plus adaptée. n'est aujourd'hui plus adaptée. Le présent amendement vise donc à adapter notre droit à ce règlement, tout en garantissant une bonne articulation entre les règles nationales, le droit des pratiques restrictives de concurrence et les nouvelles règles européennes.

: La parole est à M. le ministre délégué. La commission des finances du Sénat a amendé l'article 15 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et modifié la durée de l'habilitation accordée au Gouvernement légiférer par ordonnance afin d'assurer la transposition des directives du paquet bancaire. Les textes visant à transposer ces deux directives, notamment les ordonnances et les décrets, ont été transmis au secrétariat général du Gouvernement en vue de leur transmission au Conseil d'État. La capacité du Conseil d'État à revoir et à analyser les textes avant l'été est, à ce stade, incertaine. Or le délai de dix-huit mois fixé par la commission des finances du Sénat et prenant en référence la date d'entrée en vigueur de la loi Pacte, soit le 22 mai 2019, ferait tomber l'habilitation à légiférer par ordonnance le 22 novembre 2020, soit plus d'un mois avant le délai fixé par la transposition au 28 décembre 2020. Il est donc proposé de fixer le délai d'habilitation au 28 décembre 2020, et non en référence à un nombre de mois après l'entrée en vigueur de la loi Pacte.

les créances d'indemnité d'assurance est de nature à faire obstacle au libre choix du réparateur, désormais garanti par l'article L. 211-5-1 du code des assurances. En effet, cette interdiction oblige les assurés à avancer le coût des réparations lorsqu'ils font appel à un réparateur non agréé par l'assureur. Cette avance des frais représente une contrainte importante pour ces derniers et les incite en pratique à s'orienter vers les réparateurs agréés par leur assureur, qui bénéficient d'un système d'un système de tiers payant. Aussi, par parallélisme avec l'article 16 du projet de loi, le présent amendement vise à déclarer nulles les clauses interdisant la cession de créances à des tiers. Cela permettra aux réparateurs non agréés de dispenser les assurés de l'avance des frais, créant ainsi les conditions d'une juste concurrence

États membres d'exploiter pleinement la flexibilité prévue par les règles en matière d'aides d'État pour soutenir l'économie européenne. Cela a permis aux États membres de mettre

Plus qu'un instrument, elle en a fait un outil politique qu'elle a modifié et adapté tout au long de ces trois derniers mois, pour un montant total évalué pour l'instant par la Commission européenne à 1 900 milliards d'euros. Plus de 158

lieu, cet outil est à manier avec précaution, en raison du risque de distorsion de compétitivité entre les États membres de la zone euro. Selon la Commission européenne, il y a d'énormes différences entre les montants d'aides alloués selon les États

introduites par la directive dite « DAC 6 », transposée en droit français par l'ordonnance du 21 octobre 2019 et dont l'entrée en vigueur va être décalée par le projet de loi de finances rectificative en cours d'examen. Le mécanisme contraint les intermédiaires fiscaux, financiers ou comptables à déclarer à l'administration d'un État membre les dispositifs transfrontières potentiellement agressifs qu'ils conçoivent ou commercialisent. La directive permet aux États membres d'aménager cette obligation pour les intermédiaires couverts par le secret professionnel, le dispositif retenu par la France, comme par d'autres États membres, prévoit que l'intermédiaire doit solliciter du contribuable l'autorisation de transmettre les informations à l'administration fiscale. L'amendement vise à supprimer cette première étape en faisant du contribuable le seul responsable du respect de l'obligation de transmission de la déclaration. Une telle proposition appelle deux remarques de ma part : d'une part, j'y vois un risque que les informations ne soient pas correctement transmises à l'administration fiscale ; d'autre fiscale ; d'autre part, les risques soulevés pour le respect du secret professionnel me semblent devoir être nuancés. Il s'agit ici d'intermédiaires proposant des conseils fiscaux non liés à un contentieux. Si la profession d'avocat, en France, associe rôles extrajudiciaires et judiciaires, le dispositif concerne la phase préjudiciaire. J'estime donc qu'il est suffisamment

Sa première signataire, Mme Goulet, nous a demandé d'essayer de trouver un filtre préalable pour permettre aux avocats de respecter, si je puis dire, un certain

L'ordonnance 2020-115 constitue l'une des principales mesures nationales prises en vue de la transposition de la cinquième directive européenne anti-blanchiment, qui était l'une des priorités européennes de notre pays. Au-delà des exigences européennes de transparence financière, cette ordonnance a renforcé notre cadre national, afin de le rendre plus robuste encore à l'égard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le combat contre la criminalité financière, qu'il s'agisse du blanchiment organisé ou de terroristes cherchant à détourner des flux financiers, a toujours été et demeurera une priorité absolue et fondamentale du Gouvernement. Assurer l'intégrité de notre système économique et financier est aussi une priorité. La ratification de l'ordonnance y concourt. Les mesures que celle-ci a permis d'introduire, notamment la transparence financière des bénéficiaires effectifs, des personnes morales, des et des fiducies, sont des éléments-clés pour renforcer la robustesse de notre dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), à un moment où les criminels sont toujours présents et organisés et où la crise sanitaire expose les États à une recrudescence des risques en la matière. Ces éléments sont en outre déterminants pour la conformité aux recommandations du Groupe d'action financière de notre dispositif national de LBC-FT, qui est actuellement évalué par cette organisation. La ratification de l'ordonnance 2020-115, qui renforce notre cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, permettra de conforter la solidité de notre action et de rappeler à quel point la lutte contre la criminalité financière est notre priorité quotidienne.

en compléter le dispositif en autorisant les collectivités et leurs groupements à accorder des aides aux vétérinaires assurant des soins aux animaux d'élevage dans les zones rurales à faible densité d'élevage et caractérisées par une offre insuffisante de soins à ces animaux.

des responsabilités dans la gestion du Feader au titre du futur cadre financier pluriannuel 2021-2027, en cours de négociation. Notre point de vue n'a pas changé. Nous considérons qu'un débat

a promu, à la fin de l'année 2019, une réforme très ambitieuse, au travers du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique. Ce texte a été

Il n'a pas été retiré de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mais son calendrier d'examen demeure très incertain, pour des raisons que nous connaissons.

particulier des dispositions de la directive SMA, qui permet d'assujettir les plateformes installées à l'étranger aux obligations de financement de la production audiovisuelle et cinématographique. L'enjeu est crucial. Pendant le confinement, ces plateformes crucial. Pendant le confinement, ces plateformes ont enregistré une forte croissance de leurs revenus, tandis que ceux des chaînes de télévision, sur lesquelles repose aujourd'hui le financement de la production, subissaient les conséquences de la crise du marché publicitaire. C'est aussi le cas des dispositions de la directive relative aux droits d'auteur, qui permet de mieux protéger les droits de la propriété intellectuelle sur les plateformes de partage des contenus et de garantir le droit des auteurs et des artistes à une rémunération

à ce que les ordonnances que nous soumettrons à votre ratification respectent les équilibres nés de cette discussion. Pour le reste des dispositions du projet de loi initial,

à transposer deux directives de 2019 visant à renforcer la protection des auteurs et des titulaires de droits voisins. Ces deux directives doivent être transposées avant le 7 juin 2021. La France s'est investie de façon exemplaire dans la négociation de ces deux directives. La première renforce la capacité des titulaires de droits à être rémunérés lorsque les plateformes de partage des contenus utilisent leurs oeuvres, tout en respectant les droits et libertés des utilisateurs. La seconde stipule que les chaînes de télévision et les distributeurs sont solidairement responsables de la rémunération des auteurs

les règles concernant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias sont fixées par la loi.

Elle a fini par entraîner l'Europe dans son combat pour faire prévaloir une conception autre que celle, américaine, du. C'est en bonne partie sous l'influence française, et après un long combat, que la directive sur le droit d'auteur a pu être adoptée par le Parlement européen. Le Sénat avait d'ailleurs pesé de tout son poids, en lançant la transposition des mesures relatives aux droits voisins des éditeurs de presse avant même l'adoption finale de la directive, sur une proposition de notre collègue David Assouline.

Pour autant, il me semble que la transposition rapide de cette directive, réclamée par la quasi-totalité des acteurs de la profession, s'impose comme une nécessité aujourd'hui, au regard tant de l'incertitude du calendrier parlementaire que de l'urgence, pour les parties prenantes, de pouvoir disposer d'une vision à long terme de leur cadre de travail.

entre auteurs, artistes-interprètes, producteurs et organismes de gestion collective. Il nous revient dès lors aujourd'hui de faire un sacrifice pour donner les meilleures chances à l'ensemble d'un secteur déjà trop durement frappé par la crise,

sur ces plateformes. Il était nécessaire que l'Europe édicte des règles communes destinées à les protéger contre des contenus susceptibles de leur nuire. En France, pour les seules plateformes établies sur notre territoire, ce rôle incombera au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a su, dans le passé, protéger les auditeurs et les téléspectateurs. la France a obtenu la possibilité de soumettre à son système de soutien à la création les services qui ciblent notre territoire à partir d'autres États en dérogeant au sacro-saint principe du pays d'origine,

leur participation au financement de la création en France. L'objectif est double : d'une part, rétablir l'équité entre diffuseurs nationaux et plateformes étrangères ;

nous recherchons tous entre les services traditionnels et les nouveaux médias et à apporter des précisions sur l'association des auteurs. J'y serai évidemment tout à fait favorable. Enfin, la transposition de cette directive implique de modifier à la marge certaines dispositions de la sacro-sainte loi de 1986 qui encadre le régime de contribution à la production, pour permettre une mise en oeuvre effective des principes de la directive. créer un mécanisme de conventionnement des services à la demande pour pouvoir adapter les règles aux spécificités de chaque plateforme et de veiller à ce que les oeuvres que les plateformes déclareront au titre de leurs obligations

qui permettra la contribution des plateformes au financement de la création française, est très attendue par le monde de la création. Cette intégration à l'écosystème du financement de la création ne saurait toutefois en l'absence d'une modernisation, voire d'un assouplissement, du régime réglementaire des acteurs historiques, qui sont aujourd'hui laissés sur le bas-côté l'attente du projet de loi sur l'audiovisuel. Sans action complémentaire, les plateformes continueront à bénéficier de contraintes réduites et de droits étendus sur la production. Quant à leurs obligations de participation au financement, elles pourraient paradoxalement renforcer leur attractivité sur le marché français, grâce à des contenus premiums de qualité.

d'introduire une référence au principe d'équité entre les nouveaux acteurs et les acteurs traditionnels. Le respect de l'équité constitue d'abord une nécessité politique. Il n'est pas possible de laisser diverger de laisser diverger deux types de réglementation s'appliquant à deux catégories d'acteurs en situation de concurrence directe. Ce principe d'équité aura ensuite des conséquences juridiques,

effet, il y a des différences entre les opérateurs, mais ce principe permettra d'adapter les obligations aux spécificités respectives de chacun des acteurs. Cette rédaction, tout

pour objet d'intégrer une précision qui figurait dans le texte adopté par la commission de la culture de l'Assemblée nationale et avait recueilli un large assentiment. Il s'agit de reprendre l'interprétation du Conseil d'État concernant les modalités d'association des auteurs aux accords qui les concernent.

Nos collègues de la commission de la culture ont appelé de leurs voeux une transcription rapide de la directive SMA. La commission des finances y a été sensible et a émis un avis de

de faire contribuer les plateformes à la création et de créer les conditions d'un équilibre avec les médias traditionnels

... Cet amendement vise principalement à insérer un article additionnel habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions pour transposer la directive établissant le code des communications électroniques européen. Accessoirement, il vise à prévoir un régime de sanctions pour le règlement relatif aux services de livraison transfrontière de colis, à renforcer les pouvoirs de contrôle et d'enquête de l'Autorité de régulation des communications électroniques, à améliorer l'efficacité des procédures d'attribution de ressources en numérotation et en fréquence et à remédier à d'éventuelles erreurs du code des postes et des communications électroniques. Le choix de l'ordonnance comme vecteur législatif est adapté à la transposition d'une directive européenne technique comme le code des communications électroniques européen. Cette directive permettra de procéder à certaines adaptations de dispositions légales s'appliquant aux télécommunications spectre radioélectrique, service universel, régulation d'accès, droits des consommateurs, etc. Cette habilitation était déjà prévue dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique. Cependant, la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 qui affecte notre pays depuis mars 2020 a empêché son examen. La directive établissant le code des communications électroniques européen doit être transposée avant le 21 décembre 2020.

Le présent amendement a pour objet de transposer les dispositions relatives au service universel de la directive du 11 décembre 2018 établissant un code des communications électroniques européen. Il prévoit un cadre pour la mise en oeuvre d'un service universel au périmètre élargi, qui comprend désormais une composante relative à l'internet haut débit. Très concrètement, conformément aux exigences européennes, tous les consommateurs devront pouvoir disposer d'un accès adéquat à l'internet haut débit, ainsi que d'un système de communication vocale fixe, et ce à un tarif abordable. mesure permettra d'accéder à une liste minimale de services- messagerie électronique, presse en ligne, recherche d'emploi, etc. -fixée par le code européen des communications électroniques et qui sera codifiée par voie réglementaire. Les caractéristiques en termes de débit et de qualité de service seront également fixées par voie réglementaire en cohérence avec les objectifs arrêtés par le Gouvernement dans le cadre du plan France Très haut débit. Comme je l'ai évoqué, ces prestations de service universel devront par ailleurs être abordables. À cet égard, l'Arcep sera chargée de surveiller le niveau et l'évolution des tarifs de détail des services disponibles sur le marché, notamment au regard des prix et des revenus nationaux.

Vous le savez, l'État s'est engagé depuis plusieurs années dans le cadre du plan France Très haut débit à fournir à tous nos concitoyens un accès à internet performant à prix abordable. Le cadre juridique mis en place par le code européen des communications électroniques ne va pas modifier cet objectif ; il permet de formaliser l'objectif visé et d'imposer en cas d'insuffisance des outils de régulation et de financement déjà instaurés de nouvelles obligations aux opérateurs.

ensuite, doter d'ici à 2022 l'ensemble du territoire d'infrastructures numériques de pointe, en offrant partout un accès au très haut débit supérieur à 30 Ces objectifs, fixés en 2017, sont ambitieux, mais réalistes. Ils restent entièrement d'actualité grâce aux efforts de l'ensemble des acteurs, notamment les opérateurs télécoms et les collectivités locales, dont je tiens à saluer la mobilisation pendant la période d'état d'urgence sanitaire- cette mobilisation a permis de poursuivre les déploiements à un rythme élevé. Comme je l'ai indiqué, le cadre juridique mis en place par le code européen des communications électroniques ne va pas modifier ces objectifs.

En ce qui concerne la deuxième question, relative aux services mobiles, nous avons considéré que le Gouvernement disposait déjà des leviers nécessaires pour fixer aux opérateurs des objectifs ambitieux. L'État s'appuie pour cela sur les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui sont indispensables aux opérateurs pour fournir ces services. C'est grâce à ce mécanisme d'autorisation que le Gouvernement et l'Arcep ont pu obtenir des opérateurs mobiles, en janvier 2018, des engagements forts retranscrits depuis dans leurs autorisations en vue de généraliser une couverture mobile de qualité sur l'ensemble du territoire. Ce mobile a d'ores et déjà permis d'accélérer la couverture 4G ; il permet en particulier d'accroître la couverture des réseaux grâce à un dispositif de couverture ciblée associant l'État et les collectivités locales, mais aussi d'améliorer la couverture des axes de transport. Nous avons par ailleurs la chance de bénéficier en France d'un marché très concurrentiel avec des abonnements à très bon marché. Dans ce contexte, il ne nous semble pas nécessaire de prévoir une intervention de l'État dans ce domaine. En ce qui concerne la troisième question, un opérateur ne pourra être désigné pour fournir des prestations de service universel que s'il est établi, d'abord, qu'il existe une carence de marché, ensuite, que cette carence ne peut pas être comblée par d'autres politiques publiques comme des aides d'État, comme nous les menons en France avec le plan France Très haut débit. Le texte que nous vous proposons laisse toutes les possibilités offertes : soit une désignation nationale, soit une désignation régionale. Il permet donc de nous adapter aux besoins constatés une désignation nationale ne sera possible que s'il est démontré que la carence de marché est généralisée sur l'ensemble du territoire français. Enfin, sur la quatrième question, le Gouvernement est favorable sur le principe à ce que tous les opérateurs puissent participer, le cas échéant, au financement du service universel, y compris les opérateurs dits que vous avez cités. C'est une question d'équité concurrentielle

pour les publics les plus fragiles. Il redéfinit les obligations du service universel pour que l'accès à l'internet à un bon débit devienne un droit pour tous. Pour sa part, la le périmètre du service universel à l'accès à l'internet haut débit et donc à un ensemble de services associés. Cette directive prévoit une définition nationale du service universel, qui prend en compte le débit minimal, dont bénéficierait la majorité des consommateurs sur le territoire. Les États membres disposent du droit d'étendre le bénéfice du service universel aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises ou aux organisations à but non lucratif. Au-delà de la délimitation du périmètre de ce service universel, la France doit mettre en place un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire pour la désignation du

de la fourniture du service compte tenu de la répartition public-privé des déploiements des réseaux FTTH et de l'environnement concurrentiel, dans lequel différents acteurs déploient une boucle locale mutualisée La France retiendra-t-elle l'extension de ce service universel aux commerçants, artisans et TPE ? Quels critères seront retenus pour définir la notion de service universel abordable ? Quelles seront les caractéristiques du service d'accès adéquat à l'internet haut débit ? Comment sera défini le dispositif de réduction sociale tarifaire ? Quelle autorité assurera le suivi de la bonne application de ce tarif social et garantira le droit des usagers ? Quels seront les moyens déployés par l'État ?

Elle vise à moderniser et à simplifier le système des marques nationales et fait prévaloir la philosophie d'un système de marque au service des opérateurs économiques actifs.

se satisfont de cette ordonnance, qui apporte des changements bienvenus pour faire converger les différents droits des États membres en la matière. Dans ces conditions, la commission des affaires économiques donne un avis favorable

et d'une délibération du Conseil des ministres, lecture d'une déclaration de politique générale. Personne ne